souhaitait s'abstenir. Acte vous est donné de votre mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi rétablissant et complétant

mais il touche également à des libertés fondamentales. Il aurait donc fallu que le Sénat- lui, au moins ! -disposât de suffisamment de temps pour permettre à la démocratie délibérative de faire tout son ouvrage, dans la transparence et dans le respect

Nous avons parcouru les sentiers escarpés de ce projet de loi avec une seule idée en tête : celle du devoir, de la responsabilité. Nous avons conscience que la situation sanitaire de notre pays est grave

Ces mesures d'exception, qui donnent aux autorités sanitaires des pouvoirs exceptionnels, nous sommes prêts à les autoriser, mais non sans conditions, sans incertitude, sans inquiétude.

pensons nécessaire de prendre des initiatives fortes afin de donner un coup d'arrêt à cette flambée de la crise sanitaire. Si ce dispositif ne réussissait pas, il faudrait alors passer à des mesures plus contraignantes encore. Nous avons accepté de nous inscrire dans cette démarche. Nous avons longuement discuté avec les représentants de l'Assemblée nationale et nous sommes parvenus à un accord sur tous

des dispositifs dont le Gouvernement souhaite la mise en oeuvre, mais encore au fait que les contraintes imposées aux Français ne dépassent pas la mesure strictement nécessaire le succès de cette politique sanitaire. L'équilibre est bien difficile à trouver et- il faut avoir l'humilité de le dire -nous ne sommes pas certains de l'avoir atteint

l'esprit de responsabilité de nos compatriotes, leur conscience de la gravité des enjeux, leur volonté de protéger leurs proches et autrui et de se protéger eux-mêmes face à un risque qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, même s'il ne faut pas non plus dramatiser les choses, puisque la flambée de ce virus n'a, pour l'heure, pas été accompagnée d'une augmentation exponentielle

anticiper et agir ensemble, voilà ce que je retiens de ces jours et de ces nuits de débat

un consensus efficace, un consensus juste et un consensus qui permettra au Gouvernement, dès promulgation de la loi, après la validation du Conseil constitutionnel,

même s'il ne me revient pas d'en juger, c'est à l'issue d'un travail parlementaire extrêmement exigeant- preuve de l'attachement de chacun, sur ces travées, au juste équilibre entre nos libertés et la protection de notre santé -qu'un compromis a été trouvé entre les députés et les sénateurs, qui nous permet d'envisager, non pas sereinement,

Le passe sanitaire concernera bien les établissements recevant du public (ERP), tant en intérieur qu'en extérieur, sans notion de jauge, en incluant donc les terrasses.

devront se rendre compte que la personne ne respecte pas ou pourrait ne pas respecter les conditions d'isolement, avant de transmettre le dossier aux forces de sécurité intérieure pour qu'une intervention puisse avoir lieu, y compris au domicile de la personne

nous arrivons à un moment déterminant de la crise sanitaire. Les précédents confinements et couvre-feux se justifiaient par l'absence de vaccin et les effets insuffisants des gestes barrières. La disponibilité des vaccins et l'arrivée du variant delta changent la donne. Ce dernier représente désormais plus de 40 % des contaminations en France avec un niveau de transmission 60 % plus élevé que celui du virus original. Nous devons réaliser ce que cela représente et agir en conséquence. Actuellement, 50 % des adultes ne disposent pas encore d'un schéma complet de vaccination. Si nous maintenons le, les hôpitaux n'auront pas la capacité de faire face aux demandes d'hospitalisation, et ce dès la fin de l'été. Le vaccin protège des formes graves du virus. Se faire vacciner est non seulement un acte de protection individuelle, mais constitue surtout, ne l'oublions pas, un devoir envers la collectivité. La vaccination la plus large possible de la population est la seule priorité absolue. La question des moyens pour y parvenir a cristallisé les débats. Par les incitations qu'il crée, le passe sanitaire est une étape supplémentaire vers l'immunité collective dont la société a besoin. Notre groupe y est favorable. L'obligation vaccinale des soignants paraît indispensable pour protéger les personnes les plus vulnérables. Il n'est pas acceptable de laisser 40 % des soignants exercer au contact de personnes âgées sans cette protection. Je voudrais saluer les membres de la commission mixte paritaire, les députés et les sénateurs, qui ont trouvé le compromis indispensable à partir de positions divergentes. Nous saluons la suppression, sur l'initiative du Sénat, des possibilités de licenciement pour absence de présentation du passe sanitaire ou d'une vaccination et, sur l'initiative de l'Assemblée nationale, de l'application du passe sanitaire aux mineurs. L'extension des principes de mise à l'isolement des personnes contaminées présentes sur le territoire est une mesure importante. D'après les estimations officielles, moins de 50 % des personnes positives respectent ces mesures aujourd'hui. Nous saluons les nouvelles dispositions à cet égard. L'ensemble de ces règles s'appliquera jusqu'au 15 novembre, date qui nous paraît raisonnable. Nous devons replacer le citoyen au centre de la République. Cela passe d'abord par le respect d'un certain nombre de droits, mais aussi de devoirs. Faire société, ensemble, dans un pays démocratique, est avant tout un exercice de responsabilité. La majorité des Français est prête à faire les efforts demandés pour sortir de cette crise. Nos compatriotes s'y plient déjà depuis quinze mois avec beaucoup de bonne volonté. Ces efforts doivent être proportionnés et partagés. Le travail conjugué du Sénat et de l'Assemblée nationale a contribué à faire évoluer le texte en ce sens. La liberté est une valeur centrale pour notre groupe. Refuser délibérément de se faire vacciner, c'est prendre le risque de mettre en danger la vie d'autrui et contraindre la liberté collective. Notre contrat social repose sur une solidarité organisée. Il est temps de donner corps aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, qui font la grandeur de la France et l'honneur des Français.

Après quatre jours et quatre nuits de session parlementaire, nous terminons en urgence avec un texte qui ressemble à s'y méprendre à celui du Gouvernement. Certes, la majorité sénatoriale a obtenu la suppression des licenciements ... Ce n'est pas rien ! ... - c'était un minimum -ou la fin des mesures au 15 novembre. ou de cela, le bilan est bien maigre. Le Conseil d'État a eu plus d'influence sur la copie gouvernementale que la représentation nationale.

Au fond, la situation n'a pas changé depuis le premier confinement, où le Parlement ne siégeait pas, ou uniquement en extrême urgence pour donner les pleins pouvoirs au Gouvernement. Le covid et son corollaire d'autoritarisme technocratique sont un ultime symptôme d'une V République agonisante. Le général de Gaulle voulait remplacer le pouvoir des partis par celui des hauts fonctionnaires : « les modernisateurs », tels qu'on les appelait au lendemain de la guerre. Il a rempli son objectif dans de telles proportions que l'on imagine le résultat, soixante ans plus tard : effrayer l'homme de bon sens qu'il était. Mais gardons ce débat pour l'année prochaine, quand le Gouvernement assumera son bilan devant la France : votre bilan, c'est aussi votre méthode ! Symptomatiques de ce débat tronqué : l'utilisation de l'article 40 et votre refus de lever le moindre gage. Cela a empêché l'essentiel des débats et discussions sur d'autres propositions, exemple celle de nos collègues socialistes sur la vaccination obligatoire ou la nôtre sur un effort massif de la sécurité sociale pour informer nos concitoyennes et nos concitoyens de la nécessité de se faire vacciner. Sur ce point comme sur d'autres, vous ne nous avez pas répondu. Aussi, je vous reformule mes questions de vendredi : quand confierez-vous enfin à l'assurance maladie la charge d'une campagne massive de sensibilisation sur l'importance de la vaccination et la sécurité des vaccins ? Que prévoyez-vous pour rapprocher les plus jeunes de la vaccination ? Quelles mesures allez-vous prendre pour déployer la vaccination dans les quartiers populaires et les déserts médicaux ? Mais, surtout, pourquoi n'avoir pas déjà fait tout cela ? Si les doses manquent encore, il faut nous le dire le dire ! Votre passe sanitaire, désormais élargi aux mineurs, est encore plus injuste pour toutes celles et tous ceux qui n'étaient pas prioritaires pour se faire vacciner. On pense bien sûr à notre jeunesse, qui n'en finit pas de payer le tribut de l'épidémie et que vous ignorez d'un mépris souverain. On pense à tous les publics les plus éloignés socialement ou géographiquement de la vaccination. Plutôt que de réinstaurer des jauges dans les lieux accueillant du public, nous voilà avec cette mesure discriminatoire et liberticide. Nous avons passé l'essentiel de nos débats à parler de sanctions et de répression et pas de santé publique, le tout pour un dispositif inapplicable et inefficace qui va monter les Français les uns contre les autres et entraîner des fraudes massives. La division, le clivage, la peur du gendarme ne sont pas des méthodes que nous devrions utiliser en matière de santé publique. Voilà pour ce coup-ci, en attendant- je ne l'espère pas -le prochain variant X, mille fois plus contaminant, et la prochaine série de mesures liberticides ! Le virus continue de circuler partout dans le monde, car nous refusons, encore et toujours, la levée des brevets et de faire jouer la solidarité internationale. Apparemment, Emmanuel Macron n'a pas profité de son passage à Tokyo pour avancer sur ce sujet. Pourtant, il semble avoir eu le temps de continuer à donner des leçons aux Françaises et aux Français depuis l'autre bout du monde.

Face à un virus qui mute et dont les niveaux de contamination s'envolent, il nous faut agir. Je souhaite saluer le travail des rapporteurs, qui ont cherché à construire un texte efficace et protecteur à partir d'un constat partagé sur ces travées. Ce texte porte en lui des outils essentiels pour limiter la propagation de l'épidémie. Ils visent à assurer une protection de toute la population, tout en maintenant au maximum l'activité sociale. La liberté individuelle s'inscrit au sein d'une liberté collective que nous, parlementaires, nous nous devons de construire en garants de l'intérêt général. En l'appliquant, nous ne montons pas les Français les uns contre les autres, nous les responsabilisons. C'est tout l'objet de ce texte et de l'équilibre trouvé en CMP : une alternative à des mesures de freinage plus restrictives qu'aucun de nous n'appelle de ses voeux ; une alternative viable, surtout. Quelle autre solution assure à court terme la protection des citoyens tout en préservant au maximum l'activité de chacun, malgré la dynamique de l'épidémie ? Je n'en vois pas. Certains répondront : la vaccination obligatoire pour tous. Si l'extension de la couverture vaccinale est indispensable, plusieurs points font obstacle à la consécration de cette voie comme solution immédiate : tout d'abord, la finalisation d'un schéma vaccinal prend plusieurs semaines ; ensuite, la pédagogie doit encore primer pour les moins pour les moins enthousiastes ; enfin, l'implication de nos soignants ne fait pas de miracles, et la vaccination de tous ne se fait pas en un jour. Le passe sanitaire étendu est, à l'heure actuelle, l'outil le plus adapté. Il constitue une troisième voie, déjà approuvée par la Haute Assemblée au sein de la loi du 31 mai. La version étendue du passe est enserrée de garanties, renforcées dans la version issue de la CMP. Je veux le redire, la mise en oeuvre de cet outil reste une habilitation du Premier ministre, une capacité dont il peut se passer si la situation ne le justifie pas ou plus. Cette capacité est également encadrée dans le temps, puisqu'elle prendra fin au 15 novembre, conformément à l'accord trouvé en CMP. Je veux saluer les travaux de cette CMP. Grâce à un compromis solide, ils ont maintenu le mécanisme de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation de contrôle par l'employeur, qui paraît très adapté à la situation des ERP. Ces travaux ont également permis de revenir sur plusieurs limitations du passe sanitaire qui avaient été introduites au Sénat. Ces minorations auraient finalement privé d'effet un dispositif que les mêmes personnes considéraient comme inopérant. Le projet de loi porte également en lui une avancée unique dans la lutte contre la covid-19 : la vaccination obligatoire des professionnels de santé et de ceux qui travaillent dans des établissements au contact des personnes les plus vulnérables. Cette vaccination s'inscrit dans l'engagement qui guide leur carrière et leur devoir d'assurer la protection des plus vulnérables. Une obligation sans sanction n'a malheureusement qu'une faible portée. C'est pourquoi nous saluons le dispositif proposé pour assurer que cette obligation vaccinale soit réelle, tout en confortant son caractère transitoire pour les salariés ayant reçu une dose. Le texte présenté est à la hauteur de la situation. Avec une hausse du taux d'incidence sur tout le territoire, une augmentation des contaminations et le risque qu'elles induisent pour notre système de santé, l'heure n'est malheureusement plus aux belles idées mais aux actions fortes. Ces mesures sont proportionnées et nécessaires : le Conseil d'État, le conseil scientifique et la Haute Autorité de santé nous le rappellent. Surtout, le temps nous est compté. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera, dans sa majorité, les conclusions de la commission mixte paritaire.

fortement. J'entends les arguments selon lesquels le passe sanitaire nous priverait de notre liberté. Pour ma part, je pense au contraire qu'il peut constituer un passeport pour une liberté retrouvée, car, si nous ne prenons pas rapidement des mesures fortes, je crains qu'un nouveau confinement ne soit inévitable. Ne serait-ce pas là une bien plus grande contrainte pour nos concitoyens et un problème pour notre économie ? Cela a été rappelé, le variant delta est mille fois plus contagieux. Pour y faire face, la vaccination de masse- cela est désormais admis -peut nous permettre de gagner cette course contre la montre.

Je salue l'équilibre trouvé en commission mixte paritaire cet après-midi dans des conditions d'examen particulièrement difficiles. Je pense à l'extension du passe sanitaire aux mineurs et aux espaces extérieurs,

Nous le savons bien, si les jeunes sont beaucoup plus souvent asymptomatiques- près de deux fois plus que les adultes -, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contagieux ni transmetteurs. Je rappelle également qu'il est prévu de revoir le dispositif le 15 novembre et de l'alléger si les conditions sanitaires le permettent. L'assouplissement des sanctions à l'encontre des restaurateurs et des employés, proposé par le rapporteur de la commission des lois, va dans le bon sens, tout comme la suppression du licenciement. Je me félicite également que la CMP ait conservé la disposition proposée par notre collègue Laurence Rossignol, selon laquelle les jeunes à partir de 16 ans qui souhaitent être vaccinés contre le SARS-CoV-2, même en l'absence d'autorisation parentale, puissent le faire. C'est une excellente mesure. Les travaux de la CMP ont abouti, à mon sens, à un texte équilibré, efficace et plus protecteur, notamment grâce à l'excellent travail de nos deux rapporteurs. Pour autant, mes chers collègues, le passe sanitaire ne doit pas nous exonérer des gestes barrières, comme l'a rappelé le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, lors de son audition la semaine dernière. Il nous a expliqué combien les petits gestes allaient être fondamentaux pour notre population durant les semaines à venir. Concernant la vaccination obligatoire des soignants, là encore, j'entends bien les réticences que certains expriment. Pour autant, je souscris pleinement au principe de la vaccination obligatoire pour ces professionnels de santé. N'oublions pas qu'ils sont déjà soumis à des dispositions particulières en matière de vaccination, comme c'est le cas pour le vaccin contre l'hépatite B. Elles sont justifiées par les risques particuliers auxquels peuvent être confrontés les soignants, mais aussi par le principe de vaccination altruiste dans le but de protéger les patients.

Cet après-midi, la CMP s'est réunie et a retenu avec parcimonie un certain nombre de mesures adoptées par le Sénat. Il faut dire qu'avec son texte initial le Gouvernement avait décidé de sortir l'artillerie lourde, très lourde, en matière de restrictions des libertés publiques. Cela se voyait trop, il fallait atténuer. Les quelques modifications adoptées pourraient presque nous réjouir, car, pour certaines d'entre elles, elles atténuent effectivement des mesures plus que contestables. Néanmoins, ces modifications restent marginales et n'ont pas mis fin au passe sanitaire, même aménagé. La logique du texte gouvernemental est maintenue, comme elle l'est en matière d'atteinte au droit du travail. En effet, la suppression de la référence au licenciement introduite par le Sénat ne peut masquer le fait que les salariés concernés seront placés dans une situation statutaire et financière extrêmement difficile avec la suspension prévue de leur fonction et rémunération. Cela conduira, dans la plupart des cas, à une rupture brutale de leur contrat. Nous refusons catégoriquement l'instrumentalisation de cette crise sanitaire pour porter ainsi atteinte aux droits sociaux. En parallèle à ces sanctions salariales, les sanctions pénales ne sont pas moins insupportables. Il est question d'amendes lourdes et de peines de prison. En plus des atteintes au droit du travail, nous n'avons cessé de dénoncer des atteintes extrêmement graves aux libertés publiques, dénoncées aussi par un nombre croissant de personnes, associations et syndicats jusqu'à la Défenseure des droits et la CNIL. C'est pour cela que, dès demain, nous saisirons le Conseil constitutionnel avec le groupe socialiste du Sénat. Le Conseil jugera ainsi s'il est conforme à notre droit constitutionnel d'imposer une privation de liberté- l'isolement -sans décision de l'autorité publique, mais sur simple communication d'un pharmacien, car la majorité sénatoriale a laissé faire en CMP ; de contraindre les employés à présenter ce passe extrêmement contraignant sous peine de ne plus être rémunéré d'étendre l'accès à des données médicales et personnelles à de nombreux agents et personnels mettant en cause le secret médical ; de mettre en oeuvre un contrôle de tous par tous. Sur ce dernier sujet, l'amendement qu'a fait adopter notre groupe, qui vise à n'autoriser que les forces de l'ordre à vérifier l'identité, démontrera par l'absurde les excès insensés de ce passe sanitaire. Il est insensé, en effet, de la part du Président de la République d'avoir pris à contre-pied le peuple en passant des « jours heureux » aux « jours contraints ». Nous l'avons dit et répété, notre voie n'est pas celle de la contrainte, mais celle de la persuasion pour accélérer la campagne de vaccination et pour, un jour, en terminer avec la covid. Mais, pour cela, il faut une véritable politique de santé publique et certainement pas la société de la surveillance que vous peaufinez depuis des années, texte après texte. Ce pouvoir fracture le pays. Nous appelons, quant à nous, à l'unité face à la pandémie- unité fondée sur la confiance en nos concitoyennes et nos concitoyens -et à cesser de de les culpabiliser et de les infantiliser. Il est de la seule responsabilité du Gouvernement d'engager tous les moyens pour mobiliser et convaincre toute la société.

Lorsqu'on constate les cortèges qui gonflent jour après jour, il était important que le Sénat marque son action avec le Gouvernement.

faire face aux difficultés, en accompagnant le Gouvernement et en faisant le pari qu'il fallait, ensemble, prendre des mesures pour faire face à la maladie. C'est un pari osé, et nous espérons ne pas nous être

Monsieur le président, messieurs les ministres,

assumées comme telles. Je pense qu'il est préoccupant pour la qualité de la loi que le Parlement ne puisse travailler dans des conditions décentes. Au final,

le projet de loi. Cela permet de partager la responsabilité du mécanisme qui sera mis en place demain. Au prix de la reconnaissance d'un certain nombre de dispositions souhaitées par le Sénat, désormais,

nous nous retrouvons ce soir pour valider l'accord équilibré auquel nos deux assemblées sont parvenues, à l'issue d'une longue et âpre négociation en commission mixte paritaire. Je salue la sagesse dont ont fait preuve les membres de cette CMP, qui ont pris leurs responsabilités pour s'accorder sur les dispositifs et moyens devant permettre au Gouvernement de répondre à l'urgence que pose une reprise épidémique d'une ampleur potentiellement inédite. Je tiens à féliciter tout particulièrement notre collègue rapporteur de la commission des lois, Philippe Bas, pour la très grande qualité de son travail sur ce texte, ... Merci ! ... animé par le souci constant de concilier libertés publiques et mesures qui s'imposent pour juguler la circulation du virus.

Parmi les avancées du Sénat qui ont été maintenues et auxquelles la commission des affaires sociales a contribué figurent les assouplissements que nous avons introduits dans le calendrier et les conditions de mise en oeuvre de l'obligation vaccinale. Je pense au maintien de la période dérogatoire complémentaire du 15 septembre au 15 octobre 2021 pendant laquelle les professionnels ayant déjà reçu une dose pourront continuer à exercer leur activité, sous réserve de présenter des tests virologiques négatifs. Il s'agit de ne pas faire du 15 septembre une date couperet pour des professionnels qui se sont bien engagés dans une démarche vaccinale, mais qui, en raison d'éventuelles difficultés d'accès aux rendez-vous vaccinaux, ne justifieraient pas de l'ensemble des doses requises. La commission des affaires sociales et la commission des lois ont également veillé à assortir le non-respect de l'obligation vaccinale de sanctions proportionnées la suppression du licenciement, tiré du défaut de vaccination, constitue à cet égard une vraie victoire. Il était en effet inenvisageable de pénaliser aussi lourdement des personnes non vaccinées et de faire peser sur l'employeur le poids d'une telle décision. Nous restons convaincus que la suspension du contrat de travail devrait suffire à inciter les professionnels les plus réticents à rejoindre les rangs de leurs collègues vaccinés. Ils ont en partage une même éthique et le souci des personnes vulnérables qu'ils sont amenés à côtoyer. La commission des affaires sociales a également eu à coeur de renforcer l'expertise médicale et scientifique sur laquelle doit se fonder l'autorité publique pour prendre ses décisions dans le déploiement de l'obligation vaccinale. À l'instar de ce que le code de la santé publique prévoit pour la définition des obligations vaccinales contre l'hépatite B, par exemple, mais aussi contre d'autres pathologies, nous avons prévu que le décret encadrant les conditions de la vaccination obligatoire contre la covid-19 sera pris après avis de la Haute Autorité de santé. Il en sera également ainsi dans le cas d'une suspension de l'obligation. Il s'agit d'un élément puissant de légitimité scientifique et de sécurisation juridique des décisions qui seront prises pour mettre en oeuvre l'obligation vaccinale contre la covid. Enfin, je me félicite de l'extension du dispositif d'autorisation d'absence aux salariés ou agents publics qui devront accompagner les mineurs ou les majeurs protégés placés sous leur responsabilité à des rendez-vous vaccinaux contre la covid-19. Cette facilité n'est pas anodine, à un moment clé du développement de la couverture vaccinale de notre pays. Le conseil scientifique a en effet rappelé, au début de ce mois, que la vaccination des adolescents

paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement.

Mes chers collègues, c'est une procédure constitutionnelle non non usitée depuis plusieurs décennies qui est utilisée aujourd'hui. Après accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire,

de la déambulation dans une voie piétonne très fréquentée. C'est la raison pour laquelle nous restons fermes sur le principe pas de passe sanitaire pour l'accès aux galeries des grands complexes commerciaux. Le Gouvernement fait valoir, dans l'intérêt supérieur de la sécurité sanitaire, qu'il est nécessaire, par exception à ce principe,

Mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire. Et nous a aussi épuisés ! Je ne le sais que trop bien ... M. le président du Sénat a reçu de M. le Président de la République communication du décret portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire. Cette information sera publiée au et sur le site internet de notre assemblée. Sous réserve de la publication du décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire